adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

le rapporteur. Le présent article met en place un examen médical obligatoire préalablement au départ à la retraite de salariés ayant été confrontés à des facteurs de risques professionnels au cours de leur carrière. Cet examen médical a pour objet d'évaluer les effets de ces expositions et d'assurer leur suivi, y compris après le départ à la retraite des salariés concernés. Le présent amendement tend à codifier cette disposition au sein du code du travail ; il a reçu un avis favorable de la commission.

à la procédure qui va se mettre en place, à savoir les examens médicaux pour tous ceux qui partent à la retraite et qui peuvent, éventuellement, présenter un handicap d'au moins 10 %.

Gabouty. L'article 51 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a rendu obligatoire l'élaboration d'un plan de mobilité pour le personnel des entreprises regroupant au moins 100 travailleurs travailleurs sur un même site dans le périmètre d'un plan de déplacements urbains. Il s'agissait notamment d'encourager l'utilisation des transports en commun et du vélo, le télétravail, la flexibilité des horaires et le recours au covoiturage et à l'auto-partage. Cet amendement vise à rendre obligatoires les mesures relatives au télétravail et à la flexibilité des horaires au sein de ces plans de mobilité, les grandes entreprises ayant un rôle à jouer dans la prévention des épisodes de pollution et la fluidité des déplacements pendulaires.

Il doit comprendre un volet sur l'amélioration du transport des personnels des entreprises pour les inciter à prévoir un plan de mobilité. Ce plan de mobilité n'est obligatoire que pour les entreprises employant plus de 100 personnes. Quand ce plan existe, il peut comprendre un programme d'actions pour promouvoir les voies alternatives à la voiture individuelle, comme le télétravail. L'unique finalité de cet amendement est que ce programme d'actions comporte obligatoirement des mesures relatives au télétravail et à la flexibilité des horaires.

... Quel est l'avis du Gouvernement ?

2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective. La quatrième ordonnance prévoit notamment que le ministre du travail peut exclure de l'extension d'un accord de branche les clauses « étant de nature à porter une atteinte excessive à la libre concurrence, compte tenu des caractéristiques du marché concerné ». Cette nouvelle disposition donne donc des pouvoirs exorbitants au ministre du travail, qui se trouve placé en position d'arbitre de la libre concurrence. Le 4 octobre dernier, les routiers ont signé, au terme d'un conflit social important, un accord de branche pour permettre le maintien de diverses primes- prime de nuit, treizième mois, prime d'ancienneté. Cet accord est-il menacé

ratifie la quatrième ordonnance, n° 2017-1388, qui a apporté des adaptations au cadre juridique de l'extension et de l'élargissement des accords de branche. Cette ordonnance

qu'elles devaient contribuer à la prévention des maladies contractées au travail qui tuent régulièrement et ne font que rarement et faiblement l'objet de reconnaissance au titre des maladies professionnelles. Je vais me contenter d'évoquer les problèmes posés par le suivi lacunaire des expositions professionnelles aux pesticides. l'environnement et du travail, l'ANSES, indiquait que plus d'un million de personnes sont exposées en France aux pesticides dans le cadre de leur profession. L'Agence soulignait que de nombreuses études épidémiologiques mettaient en évidence une association entre les expositions aux pesticides et certaines pathologies chroniques. Elle citait notamment certains cancers- prostate, tumeurs cérébrales, cancers cutanés ... -, des maladies neurologiques- Parkinson, Alzheimer ... -et des troubles de la reproduction et du développement. En 2012, la mission d'information sénatoriale sur les pesticides, dont j'étais la rapporteur, constatait, quant à elle, que le système français de reconnaissance des maladies professionnelles en agriculture conduisait à la sous-déclaration et à la sous-reconnaissance massive des pathologies liées à l'exposition aux pesticides. Quelle est la cause essentielle de cette situation ? Pour les personnes malades, la documentation insuffisante de leur exposition transforme le plus souvent le processus de reconnaissance de la maladie professionnelle en parcours du combattant. Hormis pour deux pathologies inscrites au tableau des maladies professionnelles et pour lesquelles les malades bénéficient d'une présomption de causalité, se doivent de reconstituer eux-mêmes des listes d'exposition, en allant à la recherche des carnets de commandes, des factures, des vieilles étiquettes ou des bidons. Cette démarche est compliquée par l'existence d'un important temps de latence, pouvant atteindre deux à trois décennies, entre le moment de l'exposition et celui de la survenue des premiers symptômes de la maladie. Or, sans succès dans ces reconstitutions ardues et parfois impossibles, la démonstration du lien entre la maladie et la profession est d'emblée condamnée. Du côté des instances chargées d'indemniser les personnes atteintes de maladies professionnelles et accidentées du travail, l'insuffisante documentation des expositions aux pesticides entretient la faiblesse des données épidémiologiques, ainsi que des lacunes dans la connaissance scientifique et médicale des effets sur la santé de ces expositions. Ce manque de connaissances entretient la lenteur de l'actualisation des tableaux des maladies professionnelles et celle de la mise en oeuvre de mesures de protection sanitaire. Un tel rappel est utile, au moment où le Gouvernement supprime du compte pénibilité les risques chimiques, parmi

On nous dit que c'est l'expertise médicale qui décidera si les salariés doivent rester à leur poste. Pourtant, obtenir la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % équivaut, dans bien des cas, à un parcours du combattant. Quant aux autres salariés, ils partiront en bonne santé à la retraite- du moins le croiront-ils ... -, mais ils seront peut-être rattrapés, quelque temps plus tard, par le déclenchement d'une maladie. Dans ces conditions, il n'y aura ni prévention ni réparation. Voilà ce qui attend un certain nombre dont la plupart ont déjà une espérance de vie plus courte. Bref, par ces dispositions, vous allez à l'encontre du principe de justice et de lutte contre les inégalités. Or, faut-il rappeler une fois encore que les inégalités en

que le nombre de maladies professionnelles augmente de 4 % par an ou que l'espérance de vie d'une ouvrière ou d'un ouvrier soit inférieure de six années à celle d'un cadre Est-ce un signe de bien-être au travail ou de pénibilité ? Nommons les choses par leur nom, sans occulter les tristes réalités ! Ce qui n'est pas nommé n'existe pas, écrivait le psychanalyste Jacques Lacan. Alors, nommons la pénibilité

l'amendement n° 62. Le gouvernement précédent avait décidé de créer, en contrepartie de la réforme des retraites et de l'allongement de la durée de cotisation, un compte pénibilité pour les salariés ayant exercé ayant exercé des métiers pénibles, afin qu'ils puissent partir plus tôt à la retraite. Depuis 2010, le MEDEF n'a eu de cesse de tout mettre en oeuvre pour obtenir la suppression vous avez décidé de retirer la manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques des critères de ce compte.

Depuis l'entrée en vigueur du dispositif en 2015, 975 000 comptes pénibilité ont été ouverts : un tiers d'entre eux est crédité de quatre points, un autre tiers de huit. Peu de personnes sont parties à la retraite de manière anticipée, mais cela est dû aux faits que l'utilisation des points n'a été possible qu'à partir de 2016 et que les entreprises ont largement pratiqué la sous-déclaration. Le nouveau système ne permettrait que 10 000 départs anticipés à la retraite en 2018. Pourtant, les expositions à la pénibilité sont particulièrement importantes

la réparation plutôt que la prévention. Les entreprises ont obtenu la suppression de deux cotisations, alors que le choix de financement par la création d'un fonds alimenté par ces cotisations patronales traduisait la volonté d'une solidarité interprofessionnelle. Ce financement permettait aussi de responsabiliser les employeurs, en les incitant financièrement à se mobiliser : s'ils voulaient payer des cotisations moins élevées, ils devaient réduire l'exposition de leurs salariés aux facteurs de pénibilité. De plus, avec le renvoi de la mesure de l'exposition des trois critères dits ergonomiques à une visite médicale, pour pour bénéficier d'un départ anticipé, les travailleurs exposés devront s'être vu reconnaître une incapacité permanente du fait de leurs conditions de travail égale ou supérieure à 10 %, et ce sans condition spécifique quant à une durée d'exposition.

Le choix du financement par la création d'un fonds alimenté par deux cotisations patronales traduisait la solidarité interprofessionnelle, qui doit s'exercer au titre d'un risque, qui, même concentré dans certains secteurs et types d'activité, reste inhérent à l'activité économique. Il permettait aussi de responsabiliser les employeurs pour les raisons que j'ai indiquées précédemment. La cotisation de 0,01 % de la masse salariale qui finançait la C3P serait supprimée, et la branche AT-MP de la sécurité sociale, excédentaire de 900 millions d'euros en 2017, prendrait en charge les sinistres. En fait, on sort de la philosophie préventive du C3P pour revenir aux dispositions relatives à l'invalidité et à une prise en charge, non plus, mais par la sécurité sociale. Il convient de rappeler que la branche AT-MP reverse chaque année à la branche maladie 1 milliard d'euros au titre de la non-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles. Le présent amendement vise à rétablir le financement du compte personnel de prévention de la pénibilité tel qu'il était antérieurement à la publication des ordonnances. Quel est l'avis de la commission ? auteurs de cet amendement cherchent à rétablir le fonds de financement du compte personnel de prévention de la pénibilité, alimenté par deux cotisations versées par les employeurs.

considérée introduit la notion de « reconversion professionnelle » à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. Or la reconversion professionnelle a une définition très large,

des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. La caisse d'assurance maladie peut verser des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une pension d'inaptitude. La reconversion professionnelle intervient après un processus de reclassement nécessitant toujours une nouvelle formation. C'est la transformation des activités professionnelles d'un travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours de sa carrière qui doit s'adapter et changer d'activité ou de métier. Cet article signifie donc clairement que la formation nécessaire après un accident du travail ou une maladie professionnelle sera désormais prise en charge par la branche maladie, ce qui n'est manifestement pas sa mission. Quel est l'avis de la commission ? de la commission ? L'objet de cet amendement est d'interdire la prise en charge d'actions de reconversion professionnelle par la branche AT-MP. La cinquième ordonnance a prévu que les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pourront bénéficier d'un abondement de leur compte personnel de formation, qu'un décret du 29 décembre 2017 a fixé à 500 heures, pour financer une formation devant leur permettre de se reconvertir si elles ne sont plus en mesure d'exercer leur activité professionnelle. L'entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1 janvier 2019. Il s'agit

à supprimer le droit à la formation professionnelle institué par la présente ordonnance, qui constitue pourtant un progrès majeur dans la prise en charge des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ce droit à la formation qualifiante bénéficiera, à compter du 1 janvier 2019, aux victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles présentant, en raison de la gravité de leurs séquelles, un risque particulier de désinsertion professionnelle. Ce nouveau

Elle vient harmoniser l'état du droit, assurer la cohérence des textes, au sein tant du code du travail que de nombreux autres codes concernés, abroger les dispositions devenues sans objet par l'effet des ordonnances, réécrire certaines dispositions, afin d'en clarifier le vocabulaire ou d'en préciser la portée, le tout dans un souci de sécurité juridique et d'intelligibilité, et actualiser les références au code du travail dans les codes, lois et ordonnances en vigueur. Elle procède également à la correction des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d'autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la loi

Non content de nous imposer un projet de ratification des cinq ordonnances prises en septembre 2017 après des concertations éclair avec les syndicats et un passage accéléré à l'Assemblée nationale, le Gouvernement nous présente maintenant une proposition de ratification d'ordonnance par voie d'amendement. Je n'ose pas employer le mot « désinvolture » à l'égard du Parlement, même si ce terme ne suffit plus tout à fait à décrire ce comportement et ce procédé. Cette ordonnance nous est présentée comme un simple instrument de coordination juridique. la ministre, votre texte va nettement au-delà du simple cadre rédactionnel. Certaines de ses dispositions sont neutres par rapport au contenu des cinq ordonnances précédentes, mais d'autres sont plus importantes. Par exemple, vous autorisez les signataires d'un accord de branche à prévoir les conditions dans lesquelles le délai de carence entre deux CDD n'est pas applicable. Vous proposez une nouvelle définition du groupe d'entreprises, afin d'englober les groupes étrangers en matière de reclassement des salariés inaptes à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, et du périmètre d'appréciation de la cause des licenciements économiques et des reclassements. Vous supprimez l'obligation d'indiquer la finalité du prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif dans la convention entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise d'accueil. Vous donnez la primauté à l'accord d'entreprise et d'établissement sur les accords de branche étendus. là non pas des modifications rédactionnelles, mais des mesures qui affecteront négativement les conditions de vie et de travail des salariés. Il est d'autant plus grave de les glisser par voie d'amendement en fin de discussion d'un projet de loi de ratification d'autres ordonnances. Sur le fond comme sur la forme, nous voterons donc contre cet amendement

des délégués syndicaux communs au sein de la Caisse des dépôts et consignations et de réaffirmer la compétence des partenaires sociaux en son sein pour définir leurs conditions de mise en place. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Il adapte également cet article 34 aux nouvelles dispositions introduites par les ordonnances. Ainsi, il précise que la représentativité syndicale dans le groupe Caisse des dépôts et consignations est établie

La loi du 8 août 2016 a supprimé le régime des avantages individuels acquis au profit d'un maintien de la rémunération individuelle versée au salarié. Des difficultés d'interprétation rendent nécessaires des précisions quant à la mise en oeuvre de ces dispositions. Nous souhaitons préciser que ce maintien de salaire constitue une garantie de rémunération pour le salarié, au titre des seuls éléments issus de la convention ou de l'accord mis en cause ou dénoncé, et du contrat de travail. Quel est l'avis de la commission ?

La première modification porte sur les garanties définies à l'article L. 1244-2-2 du code du travail en matière de droit à la reconduction du contrat saisonnier d'une saison sur l'autre qui ont été introduites par l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017. Alors que la loi d'habilitation à l'origine de cette ordonnance prévoyait que ses dispositions ne s'appliqueraient qu'à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, l'ordonnance a introduit des modalités de reconduction de contrat de façon non supplétive. de revenir à l'esprit et à la lettre de la loi d'habilitation en donnant la priorité au dialogue social pour fixer de telles règles de reconduction de contrat. La deuxième modification précise la portée de la protection des salariés saisonniers détenteurs de mandat. Selon les dispositions actuelles du code du travail, d'une manière générale, la rupture du contrat de travail à durée déterminée, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Il en est de même, selon ces dispositions, à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement. Il est proposé de préciser que le salarié saisonnier détenteur de mandat bénéficie bien de la protection dans ces deux cas également la rupture avant le terme du CDD ; le non-respect d'une clause de reconduction prévue par contrat ou accord collectif. La troisième modification tire les conséquences de la deuxième modification en simplifiant les délais de la procédure administrative de saisine de l'inspecteur du travail pour mettre fin au contrat à durée déterminée d'un salarié détenteur d'un mandat conférant une protection.

de la commission ? Cet amendement a été rectifié postérieurement à son examen par la commission. La première partie, nouvelle, prévoit que les règles actuelles relatives au droit à la reconduction des contrats saisonniers s'appliquent à titre supplétif, à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, afin de donner la priorité au dialogue social. La deuxième partie, nouvelle également, est une mesure de simplification et de bon sens. Aujourd'hui, quand un salarié protégé voit son CDD arrivé à son terme, l'employeur doit saisir l'inspection du travail pour vérifier que la fin du contrat n'est pas entachée de discrimination liée au mandat Cette règle est trop contraignante, car elle s'applique à toutes les fins naturelles de contrat. Le présent amendement vise donc à limiter le contrôle de l'inspection du travail aux salariés protégés dont le CDD a été rompu avant son terme initial et qui n'a pas été reconduit, en dépit d'une stipulation contractuelle ou conventionnelle. La dernière partie reprend les dispositions qui étaient présentes dans l'amendement initial qu'a présenté M. Mouiller, et sur lesquelles la commission avait donné un avis favorable. Je rappelle qu'elles visent seulement à supprimer le délai d'un mois pour envoyer à l'inspection la demande d'autorisation de mettre un terme au CDD d'un salarié protégé lorsque le contrat arrive à son terme.

d'une toute petite modification rédactionnelle : au cinquième alinéa, première phrase, avant la première occurrence du mot « accord », il faudrait insérer les mots « ou par ».

qui posaient parfois problème, tout en faisant en sorte que la protection constitutionnelle des salariés détenteurs de mandat soit pleinement garantie. Le Gouvernement y est favorable.

est à M. le rapporteur. Cet amendement vise à favoriser la mobilité internationale et européenne des apprentis en s'inspirant des recommandations formulées par Jean Arthuis dans le rapport sur le développement d'Erasmus Pro, qu'il a remis à Mme la ministre du travail le 19 janvier dernier. Durant ses travaux, Jean Arthuis a identifié de nombreux freins juridiques à la mobilité des apprentis hors du territoire national et à l'accueil d'apprentis étrangers en France, du point de vue tant des obligations pesant sur les entreprises que des contraintes pédagogiques trop strictes empêchant la réalisation de ces échanges. En conséquence, il est proposé de définir un cadre incitant toutes les parties- apprentis, entreprises, centres de formation -à profiter des opportunités offertes au niveau européen par le programme Erasmus Pro. Dans la limite d'une durée d'un an, un contrat d'apprentissage pourra ainsi être exécuté à l'étranger. L'apprenti sera alors placé sous la responsabilité de son employeur ou du centre de formation dans le pays d'accueil et soumis au droit qui y est applicable en matière de rémunération, de durée du travail, de santé et de sécurité au travail, et de repos hebdomadaire. Les modalités de réalisation de cette mobilité seront formalisées dans une convention conclue entre l'apprenti, ses employeurs en France et à l'étranger, et son centre de formation. L'accueil d'apprentis étrangers en France sera facilité, puisque les dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage leur seront applicables, à l'exception de plusieurs obligations qui font aujourd'hui obstacle à leur venue en France, comme celles qui fixent à douze mois la durée minimale d'un contrat d'apprentissage ou à 400 heures par an la durée minimale de la formation et les règles encadrant les dates d'entrée en apprentissage. Il est également proposé d'élargir les possibilités de financement de la mobilité internationale des apprentis en permettant aux OPCA, de prendre en charge tout ou partie de ses coûts, notamment de vie sur place, ainsi que les cotisations sociales. Enfin, cet amendement prévoit explicitement que les centres de formation d'apprentis, les CFA, peuvent accueillir des apprentis et qu'ils doivent encourager davantage la mobilité internationale de leurs apprentis, notamment en désignant des référents dédiés à cette mission. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Chaque année, le flux est de 6 800 apprentis par an, quand plusieurs dizaines de milliers d'étudiants partent

crains que votre frilosité à l'égard de la capacité des régions à assumer l'apprentissage et à permettre des mutualisations entre des branches qui ont des moyens très

ce sujet ; il est important parce que nous avons besoin de réhabiliter l'apprentissage, qui est trop souvent décrié dans notre pays. On sait bien, pourtant, que cette forme d'insertion professionnelle

aux entreprises. Quelques minutes avant que nous reprenions la séance, je rencontrais le président et le directeur de l'Institut nautique de Bretagne, qui me rappelaient combien il était important que les jeunes qui effectuent une formation en alternance et, notamment, ceux qui ont un contrat d'apprentissage puissent

en l'assumant, parfois de manière subreptice. C'est le cas avec l'introduction, pour la première fois dans la loi, d'une définition du travail à temps partiel des personnels navigants du transport aérien comme toute durée de travail annuelle inférieure à 235 jours d'activité, sauf si un accord collectif en dispose autrement. Il apparaît que cette disposition n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les organisations syndicales intéressées ou les organisations professionnelles du secteur. En outre, eu égard au seuil légal retenu, un grand nombre de salariés du secteur deviendrait des salariés à temps partiel. De ce fait, serait ouverte une brèche dans le modèle de protection sociale et d'affiliation obligatoire de l'ensemble des navigants à la caisse de retraite des personnels navigants, ou CRPN, puisque les périodes d'inactivité sans solde liées au travail à temps alterné ne donnent pas lieu au versement de cotisations. Par ce biais, la concurrence sociale déloyale qu'entraînerait l'arrivée de nouveaux entrants pourrait fragiliser le secteur et affaiblir les droits des salariés en place. Il convient donc de supprimer cette disposition et de renvoyer la définition du travail à temps partiel des navigants à une concertation avec leurs représentants, sous l'égide du ministère des transports. Quel est l'avis du Gouvernement ?

ayant pris la mesure de la situation, je me suis engagée vis-à-vis des autorités locales, des employeurs et des salariés pour qu'on puisse

et sur la nécessité d'apporter de vraies réponses aux acteurs économiques, qui n'en attendaient pas moins. J'avais évoqué ici même combien il

mais également au nom de l'ensemble des acteurs économiques du territoire de Saint-Martin et, par extension, de Saint-Barthélemy. Je m'interdis parfois de de m'exprimer au nom de mon collègue de Saint-Barthélemy, mais je crois que le Gouvernement a fait preuve d'initiative et je saurais relayer cette

La discussion de ces 200 amendements a confirmé que, en matière de droit du travail, il y a réellement deux visions qui s'opposent. Certains voient l'entreprise comme un lieu de conflit entre salariés et employeurs, dont les relations ne seraient basées que sur un rapport de suspicion et de force. Le dialogue social ne se justifierait que pour protéger les salariés d'une menace, les employeurs ne se soucieraient que de leur profit, avec la complicité du pouvoir. D'autres, dont je fais partie, avec les membres de mon groupe et, plus largement, de la majorité sénatoriale, croient au contraire qu'il faut pouvoir avoir confiance dans l'intelligence collective de ces communautés que sont les entreprises, confiance dans la capacité qu'ont les femmes et les hommes qui y travaillent, salariés comme employeurs, à comprendre qu'ils ont des intérêts communs et qu'ils doivent agir en conséquence. Faire confiance ne signifie pas pour autant être naïf. Oui, la violence existe dans les entreprises, violence physique, violence morale, violence économique. Oui, les abus existent, chez les employeurs, chez les salariés, parfois même chez les syndicats. La violence et les abus existent dans les entreprises comme partout ailleurs. Il faut donc prévoir des garde-fous pour que les communautés dont je parlais résistent aux comportements néfastes et aux attitudes individualistes. Comme en toute chose, il y a un équilibre à trouver : c'est une centriste qui vous le dit. Je trouve pour ma part ces ordonnances équilibrées. Elles confèrent aux entreprises la souplesse nécessaire pour s'adapter, elles encouragent le dialogue entre salariés et employeurs sans pour autant renier les missions des représentants syndicaux, et elles protègent plus efficacement. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est à mes yeux un signal fort. Continuez dans cette voie, madame la ministre ! Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour aborder le second volet de votre réforme, sans doute le plus important : celui de la protection et de l'accompagnement des salariés.

donc une réelle importance pour les PME de moins de 50 employés. Il crée une possibilité de négociation par un accord collectif sans délégué syndical ; s'il y en a un, celui-ci conserve ses prérogatives. Le comité social

en cas de conflit, les indemnités prud'homales. Cela se traduira par moins de litiges et par plus d'équité sur le territoire, par plus de justice pour les salariés et plus de sécurité pour les employeurs. Dans le C3P, plusieurs facteurs étaient ingérables, notamment pour les PME. Ils ont été retirés et le C2P, le compte professionnel de prévention,

des entreprises, notamment des PME et TPE. Il faut donc que les acteurs économiques s'approprient cette réforme, qui est utile pour les salariés et qui apporte de la stabilité aux entreprises par le dialogue et le travail ensemble. Notre économie

loi. Nous regrettons le peu d'écho qu'ont eu nos débats, alors que nous nous apprêtons à voter un texte qui va profondément bouleverser le droit du travail. Comme nous avons eu l'occasion de le l'application depuis le 1 janvier de certaines dispositions des ordonnances explique certainement ce manque d'intérêt. Ces cinq ordonnances généralisent pourtant l'inversion de la hiérarchie des normes entre l'accord d'entreprise et l'accord de branche, suppriment le principe de faveur dans bien des domaines et flexibilisent le travail. Les conséquences concrètes de des travailleurs se font d'ailleurs déjà sentir dans les entreprises. La mise en place des barèmes des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, la restriction du périmètre d'appréciation de la cause économique des licenciements au territoire national, la création des ruptures conventionnelles collectives, la fusion des instances représentatives représentatives du personnel sont autant de mesures régressives qui réduisent les protections des salariés et sécurisent, parfois abusivement, les employeurs. Même si l'on peut saluer son climat serein, le débat que nous avons eu durant deux jours a confirmé le clivage que j'avais dénoncé lors de la discussion générale. Loin d'être un texte équilibré, ce projet de loi, qui s'inscrit dans le sillon tracé par la loi El Khomri, n'a aucunement été modifié, même à la marge,

développement des sciences et techniques et à leur impact sur l'organisation du travail, à la santé au travail, aux nouveaux pouvoirs des salariés dans l'entreprise pour briser la logique financière destructrice d'emplois. Nous n'en sommes pas surpris, mais nous le regrettons vivement. Pour

l'édifice que vous nous avez présenté a au moins le mérite de la cohérence. L'ennui, c'est qu'il repose sur des fondations de sable.

Il remercie également le rapporteur, ainsi que toutes les personnes qui l'ont épaulé, de la grande qualité du travail réalisé. Je ne saurais oublier l'ensemble des sénateurs présents pour la hauteur des débats et la sérénité dans laquelle ces derniers se sont déroulés.

et à la négociation et, surtout, la suppression de la généralisation des accords majoritaires, fil rouge du dialogue social. La prochaine étape sera la commission mixte paritaire. Nous croyons en un accord entre les deux assemblées, afin de continuer sur la voie du changement et de la modernité, en attendant les prochaines réformes. La

2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. La parole est